groupe socialiste et républicain, de la proposition de loi visant à rendre effectif et à renforcer le plafonnement des frais bancaires, présentée par MM. Patrick Kanner, Claude Raynal, Vincent Éblé, Mme Laurence Rossignol, M. Jacques Bigot et plusieurs de leurs collègues

en déposant cette proposition de loi au début de l'année, nous étions bien loin d'imaginer l'intensité de la crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, ainsi que les conséquences économiques et sociales dramatiques qui frappent désormais un grand nombre de nos concitoyens. si notre pays connaît une augmentation des inégalités sociales depuis plusieurs années et si la question du pouvoir d'achat est au coeur des préoccupations et du débat politique depuis 2018, la crise risque d'accentuer encore bien davantage les disparités sociales, la précarité et les difficultés financières des plus modestes. Dès lors, nous avons le devoir de définir des mécanismes visant à contenir une telle dégradation, en limitant autant que possible la baisse du pouvoir d'achat de nos concitoyens. C'est pourquoi la question des frais bancaires est si importante aujourd'hui. Ces frais maintiennent la tête sous l'eau de ceux qui sont déjà en difficulté et nuisent directement à l'efficacité des actions publiques menées pour les aider à sortir de cette situation. Ils constituent donc un levier sur lequel nous devons agir, puisque nous en avons la possibilité. C'est l'objet de la proposition de loi que j'ai l'honneur de présenter, au nom du groupe socialiste et républicain. La situation actuelle n'est plus acceptable. Ainsi, l'association 60 millions de consommateurs considérait en 2018 que les frais liés aux incidents de paiement coûtaient chaque année 34 euros en moyenne à chaque Français, mais près de 300 euros à ceux qui étaient en difficulté persistante. Cette même étude montrait aussi qu'un foyer en difficulté financière sur cinq était prélevé à hauteur de 500 euros par an au total.

sortir. Par exemple, l'aide exceptionnelle de 200 euros que le Gouvernement a mise en place pour les étudiants au mois de juin

et c'est peut-être le chiffre le plus parlant, plus de 90 % des personnes qui perçoivent moins de 1800 euros de revenus mensuels, c'est-à-dire le salaire médian en France, payent plus de 40 euros de frais pour incident par mois. Nous devons agir. Je sais que nous sommes nombreux à partager cette volonté.

À plusieurs reprises, le Gouvernement a pris des engagements ces dernières années. En réponse à la crise des gilets jaunes, le Président de la République a lui-même promis au mois de décembre 2018 de plafonner les frais bancaires pour les plus fragiles de nos concitoyens. Car, dans la crise démocratique et sociale qui venait de se déclencher avec tant de violence, l'enjeu des frais bancaires était l'une des revendications mises en avant avec force et apparaissait comme un levier sur lequel l'État pouvait agir.

; plafonner les frais d'incidents bancaires à 25 euros par mois pour les personnes aux revenus modestes n'ayant pas nécessairement besoin de l'offre. Force est de constater que ces mots n'ont toujours pas été suivis d'effets. Et pour cause : la bonne volonté du Gouvernement est moins grande que la mauvaise volonté des banques ! Ainsi, lors de l'examen du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, le Gouvernement a fait supprimer

Écoutez bien l'exposé des motifs de l'amendement de suppression déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale : « Cette disposition pourrait créer des effets d'aubaine importants ou susciter des effets indésirables, notamment en réduisant les incitations à honorer certains paiements dus. C'est de cette logique punitive qu'il faut sortir, car elle enfonce les plus fragiles et les plus pauvres et, plus largement, tous ceux dont les revenus couvrent à peine les dépenses incontournables. Même le ministre Olivier Véran a reconnu : « Je ne l'aurais pas écrit ainsi et je regrette ces mots qui n'ont pas à figurer dans un exposé sommaire quand il s'agit de frais bancaires pour des personnes précaires.

Je ne veux pas être trop long sur le dispositif lui-même. Je sais que le rapporteur, Michel Canevet, y reviendra. Je tiens d'ailleurs à le remercier de son travail au nom de la commission des finances.

atteignent au maximum le tiers du plafond général existant. Il s'agit là d'un enjeu important sur le plan social : éviter que les plus modestes ne soient ceux qui contribuent le plus en réalité, comme c'est le cas aujourd'hui. Enfin, dans la mesure où il est avéré que les établissements bancaires ne sont pas suffisamment coopératifs en matière de reconnaissance des personnes en situation de fragilité qu'ils ont toujours l'interprétation la plus restrictive possible, nous voulons ouvrir aux présidents de conseil départemental, de centre communal ou intercommunal d'action sociale, ainsi qu'à la Banque de France la possibilité d'exiger d'un établissement bancaire l'application du statut de personne en situation de fragilité. Car ce que nous constatons aujourd'hui, c'est une interprétation trop restrictive de la part des banques : certains bénéficiaires qui devraient en relever y échappent,

Les modifications suggérées permettront d'inclure les citoyens les plus durement touchés par la crise dans les dispositions que nous proposons d'adopter, comme nous l'avons déjà voté ensemble lors de l'examen du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire. J'espère que le Sénat confirmera son engagement en ce sens, comme il l'a fait, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, à une très large majorité voilà tout juste deux semaines. Mes chers collègues, l'urgence sociale nous impose de ne pas renoncer. Face à cette crise, encore plus qu'hier, nous avons le devoir de protéger les plus modestes avant les bénéfices réalisés par les banques. Sur le sujet des frais bancaires, si important pour les Français, nous avons déjà beaucoup attendu.

dans le dispositif des situations de surendettement, auquel cas elles sont automatiquement considérées comme étant en fragilité financière. Les Les établissements financiers ont aussi leurs propres critères pour définir les personnes en situation de fragilité financière, à partir du niveau de ressources ou des incidents de paiement répétitifs qui sont observés.

Cette offre spécifique, prévue par la loi depuis 2014, garantit l'accès aux services bancaires de base à un prix modique. Nous avions également fixé l'objectif d'une progression de 30 % du nombre de personnes bénéficiant de l'offre, soit environ 300 000 à l'époque. Deuxième étape, au mois de décembre 2018, nous avons élargi le principe du plafonnement à tous les clients identifiés comme fragiles financièrement, permettant à plus de 3 millions de personnes d'être éligibles au dispositif. Les banques se sont engagées auprès du Président de la République à plafonner à 25 euros par mois et à 300 euros par an les frais d'incidents bancaires pour tous les clients concernés. Ces mesures sont importantes. Elles fonctionnent aujourd'hui pour les Français touchés par la crise. Le dispositif que nous avons mis en place a démontré son efficacité pour réduire les frais d'incidents des personnes en fragilité financière.

sur cette base un bilan de l'application du plafonnement en février dernier. Il en ressort que les engagements pris par les banques en matière de plafonnement ont bien été respectés. Le plafond mensuel de 25 euros de frais d'incidents bancaires s'applique à 3,3 millions de clients. Il a permis une diminution des frais pour plus d'un million de nos de nos concitoyens. En 2019, 490 000 personnes ont bénéficié de l'offre spécifique, contre 380 000 à la fin de l'année 2017, soit une progression de plus de 100 000 personnes en quelques mois. Ces résultats sont significatifs. Sur la base de ce bilan, nous avons amélioré le dispositif pour répondre aux attentes des différentes parties prenantes. En février prenantes. En février dernier, nous avons obtenu l'engagement des grandes entreprises émettrices de factures de déployer d'ici à la fin de l'année 2021 des solutions, afin que les prélèvements infructueux représentés-

Ces entreprises vont également pouvoir proposer à leurs clients de choisir librement les dates de prélèvement pour prévenir les accidents de trésorerie. D'autres améliorations inspirées de discussions concrètes avec les acteurs de terrain vont être mises en oeuvre dans les prochaines semaines. Dans le cadre de l'examen du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, Bruno Le Maire s'est engagé à améliorer la définition de la fragilité financière, qui conditionne l'accès à l'offre bancaire spécifique et au plafonnement des frais d'incidents. Cette évolution vise à permettre aux personnes fragiles de bénéficier plus rapidement des effets du plafonnement, qui intervient aujourd'hui après trois mois. L'idée est de déclencher plus précocement ce repérage des personnes fragiles.

Cela démontre qu'il n'est pas besoin de passer par la contrainte législative pour parvenir à des résultats concrets et puissants, et que le dispositif peut être amélioré constamment en s'appuyant sur les remontées de terrain. Nous proposons donc pragmatiquement de poursuivre dans cette voie, car elle a démontré son efficacité. Au-delà de cette question de méthode, nous avons également une divergence de fond avec le dispositif proposé. Le texte de la proposition de loi

Il nous paraît difficile de défendre un plafonnement généralisé qui s'appliquerait de manière indiscriminée aux frais d'incidents et aux frais de fonctionnement normaux, lesquels rémunèrent des prestations habituelles fournies par les établissements bancaires.

Il n'y a rien d'anormal à ce qu'un client effectuant de nombreuses transactions bancaires et disposant de moyens financiers importants paye des frais, notamment en cas d'incident ; on peut effectivement estimer qu'il est suffisamment organisé pour éviter une telle situation.

à laquelle je sais votre assemblée à juste titre sensible. J'ajoute enfin que cette proposition irait à l'encontre du développement de services innovants. En effet, dans le secteur bancaire, le développement d'offres alternatives favorise le consommateur. Je pense notamment aux néo-banques, qui font partie intégrante du paysage bancaire pour nombre de nos concitoyens

En matière de frais bancaires, le dispositif de plafonnement des frais d'incidents mis en place par le Gouvernement en lien avec le secteur bancaire et les associations protège nos concitoyens touchés par la fragilité financière.

que sur les frais d'incidents bancaires. S'il me semble bienvenu de rappeler que le coût de gestion d'un incident de paiement ne se limite pas, pour la banque, au prix du timbre utilisé pour envoyer une lettre au client, est-il pour autant acceptable de constater que les citoyens les plus fragiles financièrement

à celui du modèle économique des banques dans son ensemble, notamment dans un contexte de taux bas. Si les prêts ne rapportent plus, il faut bien trouver l'argent ailleurs. Dans le retrait d'espèces

Nous avons eu l'occasion de rappeler que le taux de souscription de l'offre spécifique n'excédait pas 15 % des clients éligibles. Faut-il alors réformer le fonctionnement d'un outil considéré comme trop rigide pour ses détenteurs ? La question est posée.

Profitons dès lors de ce texte pour traduire dans la loi les engagements mis en oeuvre depuis dix-huit mois sur les frais bancaires, la loi étant par définition moins perméable aux aléas du contexte général. Le rapporteur, Michel Canevet, dont je salue une nouvelle fois le travail, propose de profiter de l'examen de ce texte pour apporter des améliorations reposant sur une logique importante, la transparence.

Mes chers collègues, je pense que l'esprit de responsabilité de Sénat peut et doit imprégner cet épineux sujet, trop souvent réduit à la caricature du banquier qui se gave sur le dos des plus modestes.

pour le groupe socialiste et républicain, la crise que nous traversons n'est pas seulement une crise sanitaire et économique ; c'est aussi une bombe sociale à fragmentation. Les mesures Les mesures prises par le Gouvernement depuis deux mois n'anticipent pas, malgré nos multiples alertes, cette situation dégradée qui attend notre pays et qui risque de s'installer pour de nombreuses années. Certes, cette proposition de loi a été pensée bien avant que nous puissions imaginer la situation actuelle. Certes, la problématique des frais bancaires est bien antérieure à la crise que nous vivons.

le dispositif que nous proposons est encore plus opportun aujourd'hui. J'ai bien entendu les remarques de M. Husson, et je sais que des amendements ne manqueront pas d'être adoptés à l'occasion de notre débat. Mais

n'accouchent que rarement d'un monde d'après plus fraternel et plus solidaire. Il nous appartient de veiller à ce que cette solidarité s'inscrive dans les faits. Si nous ne faisons rien, cette crise sera comme les autres. Les plus fragiles seront durement frappés, les inégalités augmenteront, une partie de la classe moyenne basculera dans la précarité et le populisme progressera.

pour faire face au confinement et pour accompagner le déconfinement ; des aides ponctuelles ciblées ont été débloquées. Je les salue, mais les enjeux sont bien plus larges, et le thermomètre de l'explosion de la demande alimentaire doit plus que nous alerter. Oui, l'urgence est à l'action sur le front social ! Convoquer l'esprit du Conseil national de la Résistance, comme l'a fait à plusieurs reprises le Président de la République, ne suffit pas. Il faut agir et mettre en place en urgence un nouveau pacte social national pour amortir l'effet de la crise sociale et sanitaire. Sinon, mes chers collègues, ce sont non pas des jours heureux qui nous attendent, mais des jours désastreux. Le groupe socialiste et républicain compte sur la Haute Assemblée pour engager le travail, dès maintenant, en votant cette proposition de loi, sûrement amendée. J'espère que le Gouvernement, à la lumière de ces éléments et de la dégradation de la situation sociale, se montrera plus ouvert. Qu'il cesse de qualifier d'effet d'aubaine la

Il semble donc placer la défense et la liberté d'action du secteur bancaire comme une priorité, plutôt que d'agir en direction des 80 % de nos concitoyens en situation d'endettement qui, dans les faits, ne bénéficient d'aucun plafonnement. En permettant aux banques de jouer le rôle du gendarme et, parfois, du voleur, il renforce les inégalités sociales. La situation est grave. Actuellement, près de la moitié de la population active subit une perte substantielle de ses revenus en se retrouvant au chômage partiel, et risque de rejoindre la cohorte des Français précaires asphyxiés par des frais toujours plus importants. Nous avons donc décidé que cette limitation des frais bancaires devait concerner non seulement les plus fragiles, mais également les Français qui subissent une perte de revenus temporaire en raison de la crise. Notre dispositif de limitation de ces frais permet de réguler un domaine qui ne l'est pas assez et de desserrer l'étau qui empêche de nombreuses familles de sortir la tête de l'eau pour quelques centaines d'euros. Ce n'est plus la pression des ronds-points qui doit vous pousser à agir dans ce domaine, madame la secrétaire d'État, mais la lutte contre le cataclysme social qui se dessine. Le groupe socialiste et républicain pense que la République est légitime quand elle est sociale. Ce n'est pas un effet de tribune que de le dire. Il faut regarder les choses en face. Si nous ne faisons rien, la désespérance ne sera pas seulement sociale ; elle

rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires est une démarche qui pourrait recueillir une très large adhésion au Parlement et sans doute être plébiscitée par nos compatriotes. Cette initiative relève d'une bonne intention et peut avoir son utilité dans notre réflexion sur un tel sujet. Avant de se prononcer sur ce texte, il convient de rappeler la situation du secteur bancaire et certaines caractéristiques de son fonctionnement et de son évolution. Le modèle bancaire a changé au cours de la dernière décennie, avec un produit net bancaire en légère diminution de 3 % entre 2009 et 2016 et un équilibre de ses composantes qui s'est sensiblement modifié. Si les banques se trouvent aujourd'hui parfois concurrencées par d'autres acteurs, notamment sur les moyens de paiement, leurs fondamentaux historiques- prêts, activités de marché, autrement dit les placements financiers, et commissions -résistent bien. Cependant, ils ne sont plus des vecteurs aussi dynamiques que par le passé, ce qui a conduit le secteur bancaire lui aussi à se diversifier, par exemple sur le marché de l'assurance. Cette appréciation prudente de la solidité et des perspectives de ce secteur ne nous exonère cependant pas d'examiner la pertinence des méthodes et des niveaux de frais bancaires, surtout pour ceux auxquels la loi peut conférer une base légale. Par ailleurs, il faut bien reconnaître que l'ensemble des commissions, frais, pénalités représente un vrai maquis dans lequel les clients ont souvent du mal à se retrouver et où la transparence s'affiche toujours en petits caractères. Mais avec cette proposition de loi, nous nous intéressons moins au secteur bancaire ou financier qu'à ses clients, en particulier les plus modestes, c'est-à-dire ceux qui sont souvent les plus vulnérables pour ce qui concerne la gestion de leurs revenus et de leurs dépenses. Il est vrai que ces personnes fragiles, tout comme d'autres particuliers- travailleurs indépendants, artisans, commerçants, petites et moyennes entreprises -, sont confrontées, chacune à leur niveau, aux mêmes difficultés face aux frais bancaires, ce qui peut les entraîner dans une spirale infernale pour les uns, mais profitable pour les autres. Ainsi, l'imputation des frais et pénalités du mois précédent sur un compte peut mettre celui-ci en position de découvert ou de dépassement d'autorisation, générant ainsi de nouveaux impayés

La facturation globale du découvert bancaire représentait bien 6,5 milliards d'euros de revenus en 2016, dont 4,9 milliards d'euros de bénéfices, soit 16 % du résultat net des banques françaises, qui s'élevait à

d'autre part, trop ciblée sur le public concerné. Sur le premier point, en termes de frais bancaires, il convient de bien faire la différence entre ce qui relève d'un contrat ou d'une prestation de services soumis

Il convient donc d'agir plus sur les principes et sur les pratiques que sur le montant des commissions ou des rémunérations. Sur le second point, le périmètre ne doit pas être limité au seul public en difficulté, qui bénéficie déjà des protections rappelées par Mme la secrétaire d'État, car il n'y a aucune raison que les limitations ou l'encadrement aient un caractère catégoriel, suivant des normes qui ressembleraient plus à celles d'une caisse d'allocations familiales qu'à celles d'une banque, même publique ou mutualiste. Bien évidemment, les personnes modestes, qui rencontrent, pour de multiples raisons, des difficultés, devraient être les premières bénéficiaires de nouvelles limitations ou protections, qu'il convient cependant de définir et d'adopter de manière plus générique.

Je crois cette préoccupation partagée par toutes les couleurs politiques, et je remercie mes collègues du groupe socialiste d'avoir inscrit cette proposition de loi dans le cadre de l'ordre du jour qui leur est réservé, aux termes du règlement de notre assemblée. La question, comme les choses de la vie, a toute sa place dans le débat parlementaire : les associations de consommateurs estiment à près de 6,5 milliards d'euros les frais payés par les Françaises et les Français aux établissements bancaires. Ce chiffre comporte des disparités au niveau individuel : les clients en difficulté financière persistante se voient prélever près de 300 euros de frais par an, contre huit à neuf fois moins- 34 euros -pour l'ensemble des clients en moyenne. Même si les chiffres ne sont pas objectivés faute de données fiables, les ordres de grandeur sont représentatifs de la situation des Français. Cette question a fait l'objet d'une grande attention depuis plusieurs années : depuis 2007, les tarifs bancaires liés aux incidents de paiement, c'est-à-dire le rejet par les banques d'un ordre de paiement par chèque, prélèvement ou carte, sont plafonnés, tout comme les commissions d'intervention perçues en raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire, depuis 2014. Voilà deux évolutions importantes, concrétisées sous deux majorités différentes.

En sont bénéficiaires les personnes faisant l'objet d'une procédure de traitement de surendettement, les personnes inscrites au fichier central des chèques en raison d'un chèque impayé ou d'un retrait de carte bancaire par la banque et les personnes en situation de fragilité financière selon les banques. Les mesures d'information ont également été renforcées : délai d'information avant de débiter les commissions d'intervention et présentation d'un document d'information tarifaire accessible en ligne gratuitement et distinct de la brochure tarifaire ; il s'agit de pouvoir comparer les frais bancaires d'un pays à l'autre. Les évolutions ont aussi été liées à la colère exprimée à l'occasion du mouvement des gilets jaunes en 2018. Le Président de la République s'est largement impliqué lorsqu'il a convoqué les dirigeants des principales banques et obtenu le gel des hausses des frais bancaires en 2019. D'autres engagements ont été pris, comme cela a déjà été souligné : plafonnement des frais d'incidents bancaires pour les personnes en situation de fragilité financière à 25 euros par mois, réduit à 20 euros par mois et à 200 euros par an pour les personnes bénéficiant de l'offre spécifique ; diffusion accélérée de l'offre spécifique pour la clientèle en situation de fragilité financière. Comme le note le rapporteur, Michel Canevet, dix-huit mois plus tard, force est de constater que ces engagements ont été tenus. Je ne reviendrai pas sur l'article unique de la proposition de loi, le rapporteur ayant été suffisamment précis quant aux obstacles qui doivent pousser le Sénat à amender ce texte. Les discussions entre le Gouvernement et les établissements bancaires se montrent fructueuses, sans mépris. Il me semble que les banques assument leur responsabilité dans le climat social de notre pays et répondent aux attentes toujours plus fortes et légitimes de justice. Nous croyons, en revanche, que des précisions législatives peuvent intervenir. À ce titre, mon groupe proposera deux amendements. Le premier vise à engager un effort de transparence des établissements bancaires quant aux critères qu'ils utilisent pour qualifier les personnes en situation de fragilité financière, lesquels relèvent à ce stade quasiment de leur libre appréciation. Le second repose sur le constat que la transparence permise par le document d'information tarifaire, décliné en France par application de la directive du 23 juillet 2014, n'a pas conduit à une meilleure lisibilité pour les Français, tandis que disparaît progressivement l'extrait standard des tarifs. Nous proposons donc que les banques publient dans un document unique les frais liés à douze services de base, et rien d'autre, en complément du document d'information tarifaire qui, lui, est exhaustif.

vous servir, madame la secrétaire d'État, à nourrir la réflexion sur ce sujet. Enfin, mes chers collègues, je ne peux que rappeler la complexité de ces problèmes et des transformations qui sont à l'oeuvre. La crise sanitaire a accéléré la fin de la monnaie sonnante et trébuchante des ferrailleurs de Max

Face à cette étrange affaire, il faut travailler des solutions qui, sans doute, ne relèvent pas de la loi ; je pense notamment au développement d'applications numériques européennes et sûres pour une utilisation sur smartphone. La politique est une pratique créatrice », nous dit Cornelius Castoriadis. Alors, madame la secrétaire d'abord à saluer l'initiative de mes collègues du groupe socialiste et républicain, qui nous permet de débattre en séance de la question du plafonnement des frais bancaires. Ce texte était très pertinent dès le départ ; il l'est encore davantage aujourd'hui dans le contexte que nous connaissons. Il s'agit effectivement d'un vrai sujet, dont l'origine n'est pas vraiment récente. Ainsi, une étude sérieuse, reprise par un quotidien économique sérieux il y a quelques mois, a révélé des chiffres absolument astronomiques sur l'évolution des frais bancaires. Le cabinet Sémaphore Conseil a étudié l'évolution des tarifs sur un panel représentatif de dix-huit banques depuis 2010- banques nationales, mutualistes, régionales et banques en ligne.

Ainsi, les frais de consultation de compte à distance, qui étaient encore payants pour environ 70 % des banques du panel en 2010, sont désormais gratuits partout. Dans le même temps, la gratuité des virements sur internet s'est généralisée, alors que les mêmes opérations réalisées en agence ont vu leur coût moyen augmenter de 28 %- l'étude évoque un tarif de 3,70 euros par virement. Toujours en agence, la mise à disposition de fonds coûte aujourd'hui 61 % de plus qu'il y a dix ans. Et les frais de location de coffre-fort ont progressé de 14 %, avec une facture moyenne de 99 euros. Selon cette même étude, les frais de tenue de compte sont désormais facturés, dans le panel concerné,

Les banques ne baissent pas les prix des cartes, qui restent assez coûteuses pour beaucoup d'entre elles, jusqu'à 325 euros par an pour une carte Visa Infinite en 2018, et dont les cotisations annuelles ont progressé de 5,5 % à 14,8 % sur dix ans. est le contexte général. Ces sommes pourront paraître dérisoires à des gens qui n'ont pas de difficultés en fin de mois, mais elles viennent sensiblement grever les moyens limités de nos concitoyens les plus en difficulté. Selon les associations de consommateurs, 78 % des personnes en situation d'endettement n'ont bénéficié d'aucun plafonnement et 91 % des clients touchant moins de 1 800 euros de revenus et payant plus de 40 euros de frais pour incidents par mois n'ont pas non plus bénéficié du plafonnement à 25 euros, sur lequel les banques s'étaient engagées. Par ailleurs, certains frais sont, à nos yeux, totalement injustifiés, par exemple ceux qui sont imputés lors de la saisie à tiers détenteur- c'est une véritable double peine qu'il conviendrait, selon nous, d'interdire. Citons encore le rejet de prélèvement qui est facturé 20 euros, alors que son coût administratif n'est en réalité que de quelques centimes. Autant d'opérations qui viennent alimenter le montant de 6,5 milliards d'euros cité par notre collègue dans l'exposé des motifs de la proposition de loi. Certes, la Fédération bancaire française semble contester ce chiffre,

Sans doute faudra-t-il exercer une certaine vigilance quant à l'évolution des tarifs sur l'année en cours. En effet, il faut absolument éviter une forme de rattrapage du gel de 2019. Toute augmentation serait socialement et moralement inacceptable. La force d'une loi serait la bienvenue La pandémie en cours a des effets économiques énormes ; dans ce contexte, les millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté seraient particulièrement exposés à ce risque. L'action du Gouvernement pour contrer ces effets nous semble insuffisamment volontariste et les propositions des banques souvent trop complexes, voire restreintes. C'est pourquoi le groupe CRCE est d'accord avec le présent texte qui propose un encadrement global de tous les frais bancaires. Le plafonnement proposé par ce texte permet de laisser une marge de manoeuvre assez large aux négociations entre le secteur bancaire et le Gouvernement, puisqu'il sera décidé par décret et garde la forme actuelle d'un plafonnement par mois et par opération. Toutefois, un plafonnement obligatoire par an serait, selon nous, le bienvenu. Permettre à différentes instances, comme la Banque de France ou les présidents des conseils départementaux, d'enjoindre aux banques de proposer à certaines personnes l'offre spécifique renforcerait la visibilité de cette option et du statut de fragilité financière, qui est aujourd'hui appliqué de manière plus ou moins inégalitaire selon les établissements et mériterait d'être mieux défini. La croissance soutenue des frais bancaires sur les dernières années et les stratégies de contournement des banques pour compenser les plafonnements partiels existants sont une véritable plaie sociale qui accroît les inégalités et fait des clients une variable d'ajustement pour réaliser des marges, à l'heure où les taux sont à la baisse et alors même que les banques devraient être au service Réglementer davantage le secteur bancaire incitera les banques à limiter les coûts de gestion liés aux irrégularités et les encouragera à mieux accompagner les personnes en difficulté financière. telle réglementation, nous défendons la mise en place de sanctions pour les établissements ne respectant pas les plafonnements. Des instances comme l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Observatoire de l'inclusion bancaire doivent être mobilisées pour pour aller vers plus de transparence. Nous voterons donc cette proposition de loi de bon sens qui invite à une tarification responsable et à une meilleure inclusion bancaire. La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, ce type de débat relatif aux banques est souvent l'occasion de voir se confronter deux approches. L'une présente les banques comme des acteurs incontournables au service de l'économie et les frais bancaires comme l'un des corollaires du maintien d'un réseau d'agences sur tout le territoire. L'autre verse parfois dans la critique facile d'un supposé système et dans le, les établissements bancaires étant perçus comme des machines à produire des dividendes pour les actionnaires sur le dos des clients grâce notamment aux frais bancaires.

». À propos des frais bancaires, quelle que soit leur catégorie, les citoyens les perçoivent souvent comme opaques, excessifs ou sans rapport avec le coût réel du service, bien qu'ils fassent l'objet de diverses réglementations restrictives. restrictives. Le problème existe donc bien et l'encadrement est certainement incomplet. Ces derniers mois, l'épidémie de coronavirus a causé d'importants dégâts à l'économie. Les particuliers, mais aussi les entreprises et les collectivités ont et auront besoin du soutien des banques pour traverser cette période difficile et assurer la reprise.

Après les manifestations des « gilets jaunes », l'État a obtenu des banques, en complément du gel des tarifs, le plafonnement des frais d'incident, geste que certains pourraient qualifier de timide, alors que les banques évoquent un manque à gagner significatif qui pèse sur leurs résultats. Pour autant, tout n'apparaît pas résolu, puisque le malaise subsiste entre banques et usagers. Comme pour illustrer ce dialogue de sourds, des associations de consommateurs ont relevé dans une étude publiée en 2019 que 78 % des interdits bancaires et des surendettés ne bénéficiaient d'aucun plafonnement, quand la Banque de France considère que les banques ont bien respecté leurs engagements et ont fait des progrès significatifs. Ce qui semble certain, c'est que des banques jouent davantage le jeu que d'autres, que des disparités existent entre les réseaux et les territoires, conduisant à des inégalités, et que la baisse de revenus liée au niveau très bas des taux d'intérêt conduit les banques à chercher d'autres ressources. En attendant, nombre de personnes continuent de s'enfoncer dans les difficultés, dès lors que les frais peuvent se cumuler en cas d'incidents répétés. finances, cette proposition de loi est perfectible, notamment parce que ses dispositions apparaissent à la fois trop fortes dans les restrictions qu'elles apportent et trop limitées dans leur périmètre. Néanmoins, à l'instar d'autres textes

de restaurer la confiance entre les banques et les usagers- cela me semble primordial. Nous constatons chaque jour les effets délétères d'une société de défiance citoyens mécontents, ménages en difficulté, agences bancaires vandalisées. Il nous faut avant tout sortir de cette spirale, sur laquelle prospèrent les extrêmes, et créer les conditions du rétablissement de la confiance et du dialogue. La

mais aussi de Bercy, qui souhaite laisser les banques libres d'organiser comme elles veulent la protection de qui elles veulent dans les conditions qu'elles veulent.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de loi a été déposée le 19 février dernier. Depuis, rappelons-le, la situation a beaucoup évolué au bénéfice des particuliers, notamment pour ceux qui sont les plus touchés

D'autres engagements ont été pris par les banques, comme celui de remédier à l'application répétée de frais sur un même prélèvement infructueux. Un texte devrait d'ailleurs être présenté très prochainement. Bien que pavée de bonnes intentions, cette proposition de loi me semble donc inadaptée. Faire porter le chapeau des difficultés financières de particuliers à des entreprises privées me semble contre-productif. Rappelons-le, puisque nous avons tendance à l'oublier, les banques sont des entreprises et doivent par conséquent réaliser des bénéfices. Elles doivent aussi remplir les obligations de Solvabilité 2 fixées par le législateur. Imposer à une entreprise une limitation de ses frais me semble inconstitutionnel. Je crois qu'il faut savoir raison garder et détailler un certain nombre de points fondamentaux.

Avec la baisse des taux, les bénéfices des banques de dépôt sont beaucoup plus faibles que ceux des banques d'investissement. De plus, les banques françaises subissent des pressions de la part du superviseur européen qui demande toujours plus de rentabilité par rapport aux autres modèles européens ou aux banques par internet- banques par internet- je suis pro-européen, mais j'attends autre chose de l'Europe. Revenons à notre sujet ! Chaque année, nous constatons, impuissants, des fermetures d'agences locales, des licenciements et des services de plus en plus éloignés, sans personne physique pour nous répondre. Nous pestons de voir un système bancaire qui ne peut et ne veut résoudre les problèmes non courants, comme ouvrir un compte de campagne ... En réduisant les frais bancaires, nous diminuerons les recettes et accélérerons les fermetures des agences locales dans les territoires. Est-ce cela que nous souhaitons ? Je ne le crois pas. Souhaitons-nous augmenter les licenciements et réduire l'économie sur nos territoires ? Je n'en suis pas sûr ... Au contraire, si nous voulons que les banques de proximité continuent d'exister, il faut que le législateur contribue à consolider le modèle économique des banques de dépôt. des banques de dépôt. Celles-ci veulent garder l'universalité et la relation commerciale avec tous les clients et rester des acteurs de la vie locale, quelles que soient les difficultés. Les banques sont également nécessaires pour réguler les défauts de paiement et sécuriser les échanges, en limitant les impayés par des sanctions. Il est aussi primordial qu'elles restent de proximité pour comprendre les spécificités de chaque territoire, pour connaître leurs clients. Plus cette proximité sera mise à mal, moins les banques s'intéresseront aux dossiers complexes. Avec une telle proposition de loi, j'ai le sentiment que nous déresponsabilisons une nouvelle fois les Français les plus en difficulté. Je ne suis pas sûr que ce soit générateur de situations pérennes. Demain, pour maintenir les réseaux, allons-nous les subventionner ? Il est temps de penser avant tout à ceux qui se lèvent chaque matin et qui sans cesse perdent du pouvoir d'achat, parce que la TVA, la CSG, l'impôt sur le revenu ou les taxes augmentent. Ces Français n'en peuvent plus de se sacrifier un peu plus. Ils souhaitent qu'on cesse de faire plus de social vers une minorité qui bénéficie déjà, et c'est tant mieux, de mesures très protectrices. protectrices. Vous l'aurez compris, je ne soutiendrai pas le texte proposé par le groupe socialiste, mais je m'associerai très volontiers à toutes les initiatives qui seront prises pour protéger les Français titulaires de comptes bancaires, sans mettre à mal le modèle économique des banques de dépôt. La parole

ne méritent pas d'être retenues en tant que telles. Je propose donc une réécriture générale de cet article unique non seulement pour intégrer des préoccupations permettant de faire évoluer le cadre législatif actuel, mais aussi pour répondre à un certain nombre d'interrogations qui sont ressorties des interventions des uns et des autres sur la nécessaire transparence et la clarté des informations provenant des établissements bancaires. Il importe que nous puissions analyser la situation et, pour cela,

Cela correspond aux engagements pris par la profession bancaire en décembre 2018, que nous transcrivons dans le texte. Cette mesure va permettre de protéger durablement les personnes en situation de fragilité financière contre une cascade de frais. de frais. D'autre part, il vise à assurer la transparence des critères mis en oeuvre par les banques pour identifier leurs clients fragiles

à l'heure. Tout cela est observé effectivement, cher Éric Bocquet, mais, pour ce qui concerne les clients en situation de fragilité, c'est bien l'Observatoire de l'inclusion bancaire, lequel réunit à la fois les les professionnels des établissements financiers et les organisations de consommateurs, qui constitue le lieu idoine pour appréhender cette problématique dans les meilleures conditions. Enfin, je crois que le Gouvernement s'est engagé par ailleurs à ce que

Je reviens sur ce que j'ai dit. En fait, si cet amendement de la commission était adopté, je souhaiterais qu'il soit précisé sur un certain nombre de points,

pour les banques qui l'avaient mise en place de faire en sorte que leurs clients changent de comportement lorsqu'ils avaient une tendance à se laisser aller à des irrégularités trop fréquentes. Or il se trouve que cette commission, aujourd'hui, est

L'objet de cet amendement est donc d'améliorer la transparence. Nous savons que les critères pour bénéficier de l'offre spécifique sont précisés par le code monétaire et financier : il s'agit des personnes inscrites au fichier central des chèques de la Banque de France pendant plus de trois mois consécutifs, à cause d'un chèque impayé ou d'un retrait de carte bancaire par leur banque, et des personnes faisant l'objet d'une procédure de surendettement. Néanmoins, une plus grande marge de manoeuvre est laissée aux banques s'agissant des personnes en situation de fragilité financière. Ainsi, les études réalisées par l'ACPR montrent que certains établissements bancaires usent de critères particulièrement restrictifs pour apprécier la fragilité de leurs clients. Ce sont par exemple uniquement ceux dont les revenus sont inférieurs à 1 200 euros par mois, quel que soit leur historique d'incidents de paiement. paiement. Nous proposons que les banques rendent publics, notamment sur leur site internet, le nombre de clients identifiés comme vulnérables, les critères qu'elles ont retenus et le montant moyen des frais qu'ils ont payés. payés. Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'inscrire dans la loi les engagements pris par les banques en septembre 2018, c'est-à-dire le plafonnement à 250 euros par an et à 25 euros par mois des frais bancaires pour les clients les plus fragiles, et à 20 euros par mois et à 200 euros par an pour les détenteurs de l'offre spécifique. Nous pensons en revanche

8 euros par opération et à 80 euros par mois pour l'ensemble de la population, et à 4 euros par opération et à 20 euros par mois pour les personnes bénéficiant de l'offre spécifique. je partage tout à fait l'idée de mettre l'accent sur une démarche préventive, qui est effectivement souhaitable. Simplement, le dispositif proposé risque de ne pas être opérationnel, car il est concentré sur les seules commissions d'intervention, alors même que les frais d'incident bancaire excèdent cette seule question. Les banques tendent d'ailleurs à mélanger les commissions d'intervention avec d'autres frais. frais. Il faut aussi souligner que la facturation actuelle des commissions d'intervention, lorsqu'elle est intégrée à un montant forfaitaire de frais de rejet, ne permet pas aux clients de visualiser le respect effectif du plafond. je crois que le cadre législatif actuelprévoit déjà l'information préalable du client. Le sujet relève à mon avis plutôt des modalités réglementaires de mise en oeuvre de cette information.

d'interpréter les engagements pris et, le cas échéant, de les oublier en cours de route, sur la durée. Je crois donc qu'il est important d'inscrire les obligations de transparence dans la loi. C'est ce que permet

puisque l'on a réduit le champ de cette proposition de loi par rapport à l'ambition initiale et qu'elle est tout à fait conforme à ce que voulait notre commission des finances,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, pour me conformer à nos règles déontologiques, je vais simplement dire que je suis un

Franchement, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de nous proposer, en plus de l'exemple que vous êtes en train de nous donner ? Nous devons donc être prudents, parce que l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions.

votre approche, on va poser quelques rustines pour essayer d'améliorer le système, puis on y reviendra, parce qu'on s'apercevra qu'il y a d'autres trous ailleurs qui ne sont pas supportables.

Il vise à renforcer la transparence des informations tarifaires, parce que certains établissements éditent des documents qui comportent plusieurs centaines de prix différents et, en fonction des établissements, ces tarifs sont présentés sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle. En réalité, on est face à une transparence illisible pour le consommateur, si vous me permettez cet oxymore. Pour que les consommateurs puissent plus facilement déterminer les sommes

Actuellement, les frais d'incidents bancaires ne figurent pas dans la liste des informations que les établissements de crédit ou de paiement sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public. Nous proposons de les y inclure.

l'extrait standard des tarifs qui présentait de manière synthétique les principaux frais bancaires pratiqués. Cet extrait standard reposait sur une norme de droit souple adoptée par la Fédération bancaire un argument de M. le rapporteur : il ne s'agit pas de reprendre ce que prévoit la partie réglementaire du code monétaire et financier, auquel cas notre amendement serait d'ores et déjà satisfait ; j'en ai bien conscience.

Actuellement, les établissements bancaires indiquent leurs tarifs sur une base tantôt mensuelle, tantôt trimestrielle, tantôt annuelle ; cela ne facilite pas la compréhension des tarifs et engendre des malentendus inutiles.

à ce qu'il évalue la mise en oeuvre du plafonnement des frais d'incidents bancaires appliqué aux personnes en situation de fragilité financière. Il s'agit d'assurer le suivi du mécanisme de plafonnement. À cette fin, l'Observatoire a besoin de disposer de données fiables et exhaustives sur l'ensemble des frais d'incidents bancaires. Cela permettra l'élaboration d'un diagnostic commun.

ils ne bénéficieront pas d'un dispositif qui, de fait, ne les concernera pas : cela ne coûtera donc rien aux banques. Par ailleurs, nous

dans la défense de celles et ceux qui sont le plus en difficulté. Cet amendement est très important : il est plus que symbolique, il répond à une demande très forte. Les raisons qui vous ont amenés, mes chers collègues de la majorité sénatoriale, à voter en faveur d'une disposition identique

Eh bien, je sais que la responsabilité de la situation qui nous a conduits à déposer cet amendement revient au Gouvernement, mais j'estime qu'il n'est pas trop tard, comme l'a bien

toute avancée en faveur des plus défavorisés est utile pour notre pays, dans cette période de crise sociale. Nous le ferons en responsabilité. Notre ambition était plus grande.

adresser des messages, notamment en direction du monde bancaire. Celui-ci doit comprendre qu'il lui faut aussi prendre sa part de l'effort national, dans le cadre de l'unité que nous souhaitons pour notre pays.

Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je vous rappelle que nous devrons suspendre ce débat au terme du délai de quatre heures réservé à l'espace du groupe socialiste et républicain, soit à

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, débattre aujourd'hui des conditions de la reconstruction du pacte social national dans le cadre de la sortie de la crise sanitaire, c'est aussi définir le monde d'après. Selon Jean-Jacques Rousseau, le souverain, c'est le peuple. La Constitution française témoigne que celui-ci s'est choisi une République sociale. Ce sont ces fondamentaux qui sont au principe de notre pacte social et qui doivent guider la politique qui nous permettra d'affronter la terrible crise qui se profile. Le confinement a fait apparaître les vices de notre organisation sociale et économique. Il n'a fallu que deux mois pour voir des milliers de Français basculer de la précarité dans la pauvreté ou de la pauvreté dans l'extrême pauvreté. D'ores et déjà apparaissent ceux que l'on appelle les « nouveaux vulnérables », qui représentent 4,3 millions de personnes issues des rangs des salariés les plus durement et immédiatement touchés par la crise, ceux de l'hôtellerie-restauration, de la culture, des transports entre autres.

-aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), de la réforme de l'assurance chômage. De l'alimentation au logement, la satisfaction des besoins vitaux et le respect de la dignité humaine sont des prérequis non négociables pour la septième économie mondiale. Ils n'ont pas été votre priorité. Avant la crise, vous vous glorifiiez de résultats économiques en progression, mais, au lieu d'en élargir les bénéfices, vous en profitiez pour immédiatement réduire non pas les inégalités, mais les mesures de solidarité ou de redistribution, en même temps, une politique fiscale en faveur des plus riches dans l'espoir d'un vain « ruissellement ». Comme le dit Alain Supiot, « seul le choc avec le réel peut réveiller d'un sommeil dogmatique ». Nous y sommes. Il faut réparer maintenant. Notre pacte social national doit réhabiliter quelques fondamentaux. Les premières mesures s'imposent et sonnent comme une évidence : rétablissement de l'impôt sur la fortune et de la compensation des dépenses à la sécurité sociale, restitution de leurs moyens aux associations, suppression de la réforme de l'assurance chômage ... Il faut aussi agir sur les inégalités structurelles par des politiques innovantes et commencer par la considération de ceux qui exercent les métiers dont la crise a révélé l'utilité immédiate et indispensable, ceux que certains croisent sur le quai d'une gare en disant qu'ils « ne sont rien ou ceux que les mêmes renvoient implicitement parmi les « derniers de cordée », en mettant en avant les « premiers de cordée ». Bien évidemment, la considération passe par la rémunération. Pourquoi ne pas s'intéresser à ce qui se fait au Québec depuis de très nombreuses années autour du concept d'équité salariale ? Ce principe va plus loin que le principe « à travail égal, salaire égal », puisqu'il exige un salaire égal pour un travail différent, mais équivalent. De manière générale, tous les emplois doivent être évalués à l'aune, d'une part, de leur utilité sociale, d'autre part, de quatre facteurs déterminés, qui sont les qualifications requises, les responsabilités assumées, les efforts exigés et les conditions dans lesquelles le travail est réalisé. Le résultat conduit à une augmentation sensible des salaires correspondant aux emplois d'ordinaire les plus mal payés, parce que l'utilisation de cette grille de lecture démontre à la fois la primauté de leur utilité sociale, mais aussi les conditions souvent difficiles dans lesquelles ils sont exercés. Ce concept a une autre vertu, et non des moindres, celle de donner toute leur place C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été au départ conçu. Je rappelle que les héros de la lutte contre le Covid-19 sont en majorité des héroïnes, structurellement en charge des emplois à la fois mal payés et indispensables au fonctionnement de notre société. Le personnel soignant est majoritairement féminin et huit dixièmes des vendeurs et caissiers sont des femmes, sans parler des personnels de l'aide à domicile et d'entretien. La place des femmes doit faire partie intégrante de l'évolution de notre pacte social. En France, la démarche de rémunération appropriée des professionnels est au contraire assez mal engagée. Le Gouvernement a en effet répondu à l'enjeu qui s'est imposé à la suite de cette crise par la multiplication anarchique de primes à destination de certaines des différentes catégories de personnels qui ont été en première ligne. part, ce que nous voulons, c'est au contraire très exactement ce qu'a promis le Président de la République le 13 avril dernier : que soit mieux prise en compte l'utilité sociale des métiers, pour tous, hommes et femmes. L'enjeu est de tourner le dos à la libéralisation du marché du travail et de restaurer la démocratie sociale au sein des entreprises et de la fonction publique. Pour rebâtir un pacte social qui nous convienne, l'enjeu du rapport à nos aînés est également central. personnes âgées dépendantes (Ehpad) : ce que nous y avons découvert n'est pas toujours glorieux, quand ce n'est pas carrément sordide, à l'image de ce que l'on a trouvé dans certains établissements du secteur privé lucratif. Nous attendons le contenu de vos propositions au travers d'un projet de loi relatif au grand âge et à la dépendance et nous espérons que, contrairement à d'autres projets de loi, nous serons pleinement associés dans un temps suffisamment long pour produire un travail et, à la fin, une loi de qualité. Quelles stratégies pour prévenir la dépendance ? Quelle implication du secteur public ? Comment offrir un service de prévention, puis de traitement de la dépendance égal, quels que soient les revenus ? Après la survenue de la dépendance, pourquoi ne pas imaginer des transitions plus douces et la prise en compte du lien entre les différentes générations ? Il me semble qu'il serait par exemple intéressant de réfléchir à des Ehpad intégrés au domicile. Quelles formations pour les personnels dédiés, et pas uniquement pour les personnels soignants ? La vie d'une personne âgée dépendante ne peut s'articuler seulement autour du soin et des besoins vitaux. Nombreuses sont les personnes âgées qui survivent, mais qui ne vivent plus Il est évident que toutes les générations doivent faire l'objet d'une attention spécifique. Or les plus démunis se trouvent aux deux extrémités de la pyramide des âges : les personnes âgées et les plus jeunes. Alors que nous avons eu le spectacle désespérant de résidences étudiantes devenues des zones de parcage de jeunes économiquement fragiles et n'ayant pas nécessairement les moyens de se nourrir, la mise en place d'un revenu de base d'un montant suffisant s'impose comme une nécessité, pour les jeunes comme pour d'autres. Un nombre croissant de jeunes sont laissés sur le côté pour de multiples raisons, dont la transmission intergénérationnelle de la pauvreté, avec un ascenseur social en panne et une éducation nationale qui, malgré l'implication et le dévouement de ses personnels, ne parvient pas à briser le mur séparant enfants issus d'une famille au capital socioculturel élevé et ceux qui sont pourvus d'autres richesses. Il faut casser à la base la spirale infernale du déterminisme social. Cela passe, nous le savons tous, par des politiques d'accompagnement dès la petite enfance par l'amélioration perpétuelle des dispositifs en faveur des jeunes tels que la garantie jeunes mise en place sous le quinquennat précédent, qui a fait largement ses preuves et dont il va falloir ouvrir les vannes pour aider les primo-demandeurs d'emploi dès maintenant. Nous savons en effet que la génération des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi cette année sera la première sacrifiée. Je ne peux bien évidemment pas ici brosser le tableau de tout ce qu'il est nécessaire de mettre en place dès aujourd'hui pour que n'explose pas notre vivre ensemble à la sortie de cette crise. Je conclus en rappelant que la redéfinition de notre pacte social national doit faire coexister dans l'harmonie les différentes composantes de notre société, en assurant toujours plus de justice entre classes sociales et générations.

je remercie le groupe socialiste et républicain d'avoir inscrit à l'ordre du jour de la Haute Assemblée un débat sur notre pacte social et sur les mesures nécessaires pour le renforcer dans la période de sortie de crise sanitaire. Avant d'envisager les évolutions futures de ce pacte qui nous unit, permettez-moi de revenir sur le rôle essentiel du pacte social français dans les dernières semaines. Je l'ai souvent répété : nous avons eu de la chance de ne pas avoir dû improviser un système de protection sociale dans l'urgence de la crise. Le filet de protection que nous avons tendu pour protéger les Français des conséquences de l'épidémie a joué pleinement son rôle. Nous avons tout d'abord maintenu les revenus des travailleurs en mettant en place un dispositif d'activité partielle massif qui, au plus fort de la crise, a touché plus de 12 millions de salariés. La protection sociale complémentaire a également été maintenue pour l'ensemble des salariés. Nous avons créé un dispositif d'activité partielle dédié pour les particuliers employeurs, qui a notamment bénéficié aux assistants maternels, dont l'activité était particulièrement affectée. Nous avons versé des indemnités journalières à tous ceux qui devaient cesser leur activité, parce qu'ils présentaient une vulnérabilité particulière à l'égard du Covid-19 ou parce qu'ils devaient garder leurs enfants. Nous avons veillé à éviter toute rupture de droits en rendant automatique le versement des minima sociaux pour tous les bénéficiaires empêchés de faire leur déclaration pendant la période épidémique. Nous avons travaillé avec les collectivités locales, avec les acteurs du champ social et médico-social, avec l'ensemble des services de l'État pour que, partout sur notre territoire, chacun puisse voir ses besoins essentiels Nous avons en particulier travaillé au maintien de l'aide alimentaire. Nous avons constitué une réserve sociale et une réserve civique pour soutenir les associations en manque de bénévoles. Nous avons demandé aux préfets de coordonner la poursuite des distributions, département par département, pour que les associations soient accompagnées dans la mise en oeuvre des gestes barrières, pour que des locaux municipaux adaptés au contexte sanitaire soient mis à disposition, que les bénévoles puissent se déplacer et que les nouveaux dons alimentaires parviennent bien aux associations. Nous avons mis en place un plan d'urgence d'aide alimentaire à hauteur de 39 millions d'euros, pour soutenir les associations à hauteur de 25 millions d'euros, d'une part, pour apporter une aide d'urgence alimentaire aux territoires en souffrance à hauteur de 14 millions d'euros, En parallèle, nous nous sommes très fortement mobilisés pour maintenir le service public de l'hébergement. La trêve hivernale a été prolongée jusqu'au 10 juillet prochain. Des centres spécialisés pour sans-abri atteints de formes non graves du Covid-19 ont été ouverts sur l'ensemble de notre territoire de nombreuses places d'hébergement ont été mobilisées par l'État dans des hôtels, dans des établissements publics, dans des bâtiments vacants. Au total, 178 000 places d'hébergement d'urgence sont ouvertes tous les jours et financées par l'État, contre 157 000 avant le début de la crise sanitaire. Pour compléter ce dispositif, nous avons décidé de verser une aide exceptionnelle de solidarité aux ménages les plus en difficulté. Cette aide a été versée automatiquement le 15 mai dernier à 4,1 millions de foyers sans qu'aucune démarche soit nécessaire de la part des bénéficiaires. Nous avons également souhaité apporter un soutien spécifique aux jeunes âgés de 18 à 25 ans, dont certains se sont retrouvés dans des situations de grande précarité. Une aide de 200 euros sera versée à 800 000 d'entre eux prochainement. C'est à mes yeux un enseignement majeur de cette crise : la solidarité nationale, socle de notre pacte social, a joué pleinement son rôle. Toutefois, cette crise cette crise a également mis en valeur certaines failles de notre système de protection sociale et nous devons aujourd'hui consacrer tous nos efforts à les combler plutôt que reconstruire ou renforcer notre pacte social national. Le constat de la pauvreté en France ne date pas de cette crise. Nous l'avons dressé dès notre arrivée au pouvoir et nous avons engagé des chantiers et des moyens inédits pour la faire reculer. Je pense tout d'abord à la stratégie de lutte contre la pauvreté, qui mobilise 8,5 milliards d'euros pour faire de l'investissement social et donner aux structures qui accompagnent les plus fragiles au quotidien les moyens de les extraire de la pauvreté. Je pense à l'augmentation des prestations et ressources financières de nos concitoyens les plus fragiles, avec la revalorisation de 100 euros par mois de l'allocation aux adultes handicapés et du minimum vieillesse, et à l'augmentation massive de la prime d'activité qui touche les travailleurs précaires. Je pense à la complémentaire santé solidaire ou au dispositif « 100 % santé » mis en place pour que nos concitoyens les plus modestes n'aient plus à renoncer à se faire soigner. Ce ne sont que quelques-uns des chantiers que nous avons engagés et que nous devons aujourd'hui plus avant. C'est tout l'enjeu du plan de sortie de crise sur lequel travaille actuellement le Gouvernement. Ces travaux ne sont pas achevés, mais je souhaite aujourd'hui vous faire part des trois axes qui me semblent les plus essentiels pour renforcer notre pacte social. Le premier axe consiste à garantir à chacun la possibilité de répondre à ses besoins essentiels. Je pense en particulier à la simplification de l'accès au droit et à la lutte contre le non-recours, ce qui implique notamment de développer davantage l'offre de domiciliation, les démarches d'« aller vers » des organismes de sécurité sociale. Je pense également au déploiement d'une politique publique de lutte contre la précarité alimentaire de nature à absorber la hausse des besoins engendrés par cette crise. Il s'agit de sécuriser les financements et les approvisionnements des opérateurs, de renforcer le maillage territorial, d'étendre la tarification sociale des cantines et la distribution des petits déjeuners à de nouveaux territoires, d'articuler la politique de lutte contre la précarité alimentaire avec celle de l'insertion par l'activité économique. Je pense à l'accès aux soins des plus fragiles, que nous devrons renforcer encore en articulant mieux les missions des acteurs sanitaires et sociaux, en augmentant les moyens humains et financiers permettant d'aller vers les publics vulnérables, en renforçant les permanences d'accès aux soins mobiles, les maraudes médicalisées.

Le deuxième axe essentiel est le soutien au pouvoir d'achat des ménages et le maintien ou le retour à l'emploi. Je l'ai dit, nous avons décidé la semaine dernière de verser des aides financières exceptionnelles pour soutenir les publics les plus vulnérables, dans un contexte particulier. Nous devrons tirer tous les enseignements de cette période afin que nos prestations soient plus réactives et équitables et qu'elles permettent de lutter davantage contre le non-recours aux droits. Nous devrons aussi nous donner les moyens de faire face aux conséquences de la crise sanitaire sur le marché du travail en renforçant tout particulièrement l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi et en accordant une attention spécifique aux secteurs les plus durement touchés. Nous devrons continuer à lever les freins à l'emploi contre lesquels nous luttons depuis bientôt trois ans, développer l'accès aux modes de garde, accélérer le déploiement des crèches à vocation d'insertion professionnelle. Pour terminer, le troisième axe doit concerner les jeunes, en particulier dans les territoires les plus fragiles. C'est l'un des principaux constats qui nous a conduits à concevoir la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Le taux de chômage des jeunes demeure trop élevé. La France compte 60 000 mineurs

En France, ce pacte garantit un droit fondamental : l'accès à la santé pour tous. Mais la présente crise sanitaire, et les nombreux appels des professionnels de santé qui l'ont précédée, ont durement démontré la nécessité d'une réforme d'ampleur.

Il faut bien évidemment revaloriser les salaires. Un médecin généraliste allemand gagne plus de quatre fois le salaire moyen de son pays, contre 2,9 fois pour un médecin français. Le salaire moyen des infirmiers français est l'un des plus faibles des pays de l'OCDE. Ces revalorisations devront viser les métiers paramédicaux, mais également l'ensemble des personnels hospitaliers. Il est également impératif de revoir les statuts des personnels. En effet, les professionnels et les services de santé sont étranglés par les rigidités d'une fonction publique qui n'accorde aucune souplesse. Il faut valoriser les carrières, renforcer l'attractivité des hôpitaux, qui peinent à recruter et à fidéliser leurs salariés, et pour cela revoir leurs conditions de travail. Il faut s'attaquer à la « suradministration » du système de santé et donner plus de poids aux médecins. Le fonctionnement des hôpitaux privés est éclairant. L'hôpital public a aujourd'hui besoin d'autonomie, il doit pouvoir choisir ses praticiens, adapter les rémunérations, les heures supplémentaires, le choix des équipements, l'organisation des services. Un débat sur la gouvernance Il s'agit de réformes structurelles ; partagez-vous cette ambition, madame la secrétaire de l'ensemble des professionnels de santé, dans les cabinets de ville, mais aussi dans les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. Notre système de santé a été mis à rude épreuve. Pourtant, il a tenu et s'est montré réactif, agile et d'une résilience sans pareil. Nous avons vu des professionnels de santé s'organiser pour mettre en place des parcours de prise en charge rapide des patients atteints du Covid-19 ou susceptibles de l'être. Je tiens également à saluer le rôle majeur qu'ont joué les infirmiers libéraux dans la continuité de la prise en charge à domicile, dans des conditions souvent difficiles, notamment auprès

Requier. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord remercier nos collègues du groupe socialiste et républicain d'avoir engagé ce débat qui nous impose de réfléchir aux moyens que nous souhaitons mettre en oeuvre pour soutenir les plus vulnérables. La violence de la crise sanitaire et le confinement auront en effet mis en évidence la précarité de plusieurs millions de nos concitoyens et accentué une partie des inégalités existant au sein de notre société. Je pense tout particulièrement aux jeunes,

quand survient une crise économique. Pour les plus précaires, le Premier ministre a annoncé le 4 mai dernier devant notre assemblée une aide spécifique de 200 euros, laquelle concernera 800 000 jeunes et étudiants en difficulté. Si l'on peut bien évidemment se féliciter de cette mesure ponctuelle, il nous paraît nécessaire d'activer d'autres leviers. Dernièrement, plusieurs voix se sont élevées pour demander l'ouverture du revenu de solidarité active aux moins de 25 ans,

Il évoque en revanche l'idée d'introduire des mesures pour l'emploi des jeunes dans le plan de relance prévu pour la rentrée. Madame la secrétaire d'État, ma question est simple : quelles sont les différentes pistes envisagées par le Gouvernement pour que nos jeunes ne soient pas la « génération sacrifiée du coronavirus »

La crise qui a endeuillé la France nous a contraints à nous recentrer sur l'essentiel : la santé, la famille, la solidarité. Elle a permis de faire renaître la solidarité de tous les jours, comme en témoigne le fait que 300 000 Français aient rejoint la réserve civique la plateforme jeveuxaider.gouv.fr. Force est de constater que cette crise, comme les précédentes, qu'elles aient été sociales, économiques ou sociétales, ont montré que les croyances ont évolué, mais surtout que les attentes des citoyens envers la puissance publique, notamment en pareille période, sont très C'est pourquoi il est urgent de reconstruire le pacte social, qui est au coeur des solidarités collectives, tout en stimulant les solidarités individuelles mises en lumière par la crise. Ce que révèle déjà cette pandémie, c'est que « la santé gratuite [ ...], notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe », pour reprendre les propos du Président de la République lors de son allocution du 12 mars dernier. Notre protection sociale, c'est ce qui nous permet de faire société. Hier, le ministre des solidarités et de la santé a annoncé la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale, telle qu'elle a été pensée en 1945. Attendu

À titre d'exemple, j'évoquerai la contractualisation entre l'État et les départements dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Cette contractualisation permet d'octroyer des moyens supplémentaires aux départements afin qu'ils puissent réinvestir le champ de l'accompagnement et de l'insertion sociale, notamment des bénéficiaires du RSA,

Il est donc nécessaire, voire d'une urgence absolue, de changer de logiciel. On voit où la loi du marché nous a conduits ! Elle a provoqué un affaiblissement de l'hôpital et du système de santé, quitte à mettre en danger l'ensemble de la population, mais aussi de tous les services publics qui structurent la solidarité nationale. Elle a ensuite mis à genoux le coeur de l'économie notre industrie. Tout démontre que l'argent a pris le dessus sur l'intérêt général. L'argent roi est bien la clé d'un nouveau contrat social. Une nouvelle répartition des richesses est la voie

beaucoup plus loin ! Supprimons les dispositions qui protègent de manière éhontée le capital, comme la ; agissons de manière déterminée contre l'évasion fiscale ; ramenons l'échelle des salaires à un écart raisonnable de un à vingt ; construisons un pôle public bancaire et financier pour donner à l'État les moyens d'agir et de se dégager

le retour des investissements dans notre pays. Je le répète, l'impôt n'est pas la réponse, d'autant que, comme le montrent les dépenses que nous avons engagées, l'État prend entièrement ses responsabilités pour faire vivre la solidarité nationale.

Madame la secrétaire d'État, la crise a révélé les vulnérabilités de notre modèle social, mais également ses forces adaptatives, comme un catalyseur d'évolutions prêtes à émerger. Ce phénomène est flagrant dans le domaine du travail. Entre mars et mai 2020, des millions de salariés ont poursuivi leur activité à distance. Si les grèves provoquées par la réforme des retraites ont été une sorte de répétition générale, il semble que l'épidémie de Covid-19 bouleverse durablement notre modèle traditionnel d'organisation du travail. À l'aune de cette expérience à marche forcée, 62 % des Français plébiscitent le recours au télétravail. Si certaines entreprises annoncent vouloir recruter des télétravailleurs à temps complet, d'autres proposent un modèle hybride.

En effet, l'enjeu sous-jacent est celui de l'égalité territoriale : 75 % des salariés intéressés par un télétravail à temps complet envisageraient de déménager. Cela nous conduit à considérer le télétravail comme un moyen de désengorger les centres urbains surpeuplés et pollués, où les loyers sont hors de prix. Il est donc un moyen d'offrir à la France une nouvelle politique d'aménagement de son territoire. Dans cette perspective, un cadre national est indispensable afin d'éviter que la généralisation du télétravail ne se traduise par une délocalisation des emplois qualifiés vers des pays à bas salaires.

du dialogue social et, bien évidemment, de la solidarité. Je limiterai mon propos à l'amélioration du pouvoir d'achat. Plusieurs pistes peuvent être étudiées. La généralisation de l'intéressement peut être une des voies de relance après la crise sanitaire. Il existe déjà des plans d'intéressement dans les entreprises, mais cet outil est sous-utilisé. Relançons-le en l'améliorant. Une telle mesure ne coûterait pas un euro aux finances publiques et associerait pleinement chaque salarié au redressement du pays. Autre piste : le projet de loi sur les retraites. Le Gouvernement a décidé de surseoir à son examen. Néanmoins, un certain nombre d'avancées sociales avaient été actées : le minimum retraite, la lutte contre les effets pervers des carrières hachées, notamment pour les femmes, et la revalorisation des retraites des agriculteurs.

Pourquoi ne pas expérimenter cette mesure afin de lutter notamment contre la précarité des plus jeunes et soutenir les ménages les plus pauvres et les travailleurs les plus fragiles ? ? Madame la secrétaire d'État, je crois que ne pas transformer notre modèle social serait une erreur historique. Pour réussir, il faudra, à l'instar de ce que proclamait Danton en 1792 : « De l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace ! » La parole est à Mme la secrétaire

Ce texte comporte une série de mesures qui visent à inciter les entreprises à mettre en oeuvre des accords d'intéressement. Je pense notamment à la suppression du forfait social sur l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés et sur la participation pour les entreprises de moins de 50 salariés. La loi Pacte prévoit également des accords d'intéressement types négociés types négociés au niveau de la branche et adaptés aux secteurs d'activité pour faciliter leur déploiement dans les petites et moyennes entreprises. Il s'agit de mesures qui vont dans le bon sens et que vous défendez. En ce qui concerne vos interrogations

L'apprentissage est également en danger. J'ai la conviction que cette filière d'excellence doit être soutenue. Dans la réflexion sur le pacte social, il est indispensable de consacrer un volet de soutien à l'apprentissage,

Mais l'entrée en apprentissage s'annonce fortement impactée : les prévisions de baisse du nombre de contrats en apprentissage se situent entre 30 % et 50 %. En effet, les entreprises, fragilisées par la baisse d'activité, vont être très frileuses pour recruter des apprentis. Cette baisse va elle-même entraîner un problème de financement des centres de formation : c'est un cercle infernal qui va entraîner des fermetures de classes et,, un risque de disparition de compétences pour les métiers. Vous le comprenez, l'apprentissage est en danger. Les régions ont fait la preuve de leur agilité et de leur réactivité lorsqu'elles exerçaient cette compétence, mais vous avez souhaité modifier cette gestion. cette transition va être difficile, notamment à cause des lourdeurs administratives. Il me semble donc aujourd'hui nécessaire de sécuriser les parcours des apprentis,

des outils pour accompagner les entreprises qui feront le choix de recruter et de maintenir des apprentis. Il faut envisager, par exemple, d'allonger la durée du statut de scolaire alternant aux candidats à l'apprentissage qui ne parviendraient pas à trouver

La crise a eu un impact particulier sur les précaires, ce qui pose de manière indiscutable la question de notre système de soutien aux revenus des plus précaires. J'ai

Henno. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le confinement mis en place pour lutter contre le développement du Covid-19 restera une période dont il faudra longtemps pour mesurer les conséquences sanitaires, mais aussi économiques et sociales.

L'organisation de nos travaux a changé depuis maintenant plusieurs semaines, dans des proportions que nous n'aurions jamais imaginées jusqu'ici. Le phénomène du télétravail modifie et va modifier en profondeur notre manière d'appréhender nos vies et aura un impact significatif. Les atouts du télétravail sont nombreux : gain de temps, économie d'espace et de transport- ce qui est appréciable en cette période si particulière -, meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle,

de nombreuses conséquences sociales en termes de management, avec des risques d'isolement, en termes de relations sociales et de construction d'un projet collectif d'entreprise, mais aussi de représentation des salariés. Il représente une mutation profonde et accélérée de notre environnement économique et social. Madame la secrétaire d'État, comment voyez-vous l'évolution du paritarisme et du dialogue social dans ces conditions ? N'est-il pas l'heure d'organiser une grande conférence sociale et, pourquoi pas, de proposer de nouvelles lois sociales refondées afin d'aborder, dans le dialogue social, ces mutations profondes ? La parole

de la République avait annoncé une série de mesures prises en réponse à la crise des « gilets jaunes » et tenant compte des résultats du grand débat national. La mise en oeuvre de ces mesures a été freinée par la crise sanitaire. Il faut désormais les réinvestir politiquement, les faire mûrir et les évaluer. Tout le monde a subi cette crise. Ce fut un choc symétrique. Certains, il est vrai, l'ont subi plus fortement que d'autres. Mais il ne s'agit pas de prévoir une aide financière conjoncturelle en une seule fois. Il faut envisager la reconstruction sur le long terme, aux côtés des institutions et des entreprises. Ce nouveau paradigme de société passe par trois points : l'alliance des secteurs public et privé pour l'intérêt général, la solidarité entre Français et l'implication de nos collectivités territoriales. Sur ce dernier point, les mesures du Gouvernement doivent nécessairement être le fruit des remontées du terrain, avec les maires comme premiers interlocuteurs qui enrichissent la réflexion à l'échelle nationale. À l'échelon local, il devient nécessaire de créer une cellule de veille sanitaire et sociale. Madame la secrétaire d'État, après le grand débat et cette crise sans précédent, quels outils comptez-vous mettre en place auprès des collectivités territoriales pour faire face, de manière pérenne, aux risques sociaux et sanitaires ? C'est une question que beaucoup d'élus se posent. La parole est

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le confinement a rendu visible ce que vous ne voulez pas voir : la précarité des travailleurs « ubérisés », dépendants des plateformes de livraison, et les chauffeurs de VTC, dont le droit dit

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, crise financière, crise écologique, crise démocratique et aujourd'hui crise sanitaire : nous sommes bien devant une crise durable. D'un côté, les plus forts d'entre entre nous, une minorité très qualifiée, de mieux en mieux payée ou vivant de la spéculation et non du travail de l'autre, les plus faibles qui fournissent, dans le meilleur des cas, des biens et des services locaux ou qui vivent de l'assistance apportée par l'État-providence. Entre les deux, une solidarité qui s'effrite inexorablement. L'addition est lourde mécontentement généralisé des citoyens vis-à-vis de la démocratie représentative, accusée d'être impuissante ; sécession sociale et morale des élites ; sécession territoriale des pays ou régions les plus riches. Mais voilà qu'aujourd'hui tout doit être sacrifié sur l'autel du sacro-saint pragmatisme il n'est plus nécessaire de parlementer indéfiniment pour savoir si une politique est bonne ou mauvaise, il faut seulement savoir si elle est efficace ou non. Une fois cela posé, il n'y a plus de débat idéologique possible, mais seulement des questions techniques qui ne qui ne concernent alors plus les citoyens, mais les experts, ceux qui savent comment fonctionne la machine d'État. Ainsi la démocratie s'achève-t-elle en technocratie. Nous y sommes précisément L'heure n'est plus au bricolage et à l'accumulation de dispositifs incompréhensibles. Il est maintenant extrêmement urgent de définir enfin ce que nous considérons comme une priorité à respecter, une ressource à préserver et comme un bien à conserver. Dans ce contexte, réhabiliter la Nation peut paraître contre-intuitif aux bonnes consciences humanistes, progressistes, sociales-démocrates, écologistes, et j'en passe ... Il nous faut pourtant non seulement réhabiliter la Nation, mais la réinventer. Nous devons redéfinir le pacte social national afin de le mettre tout entier au service d'une pratique sobre et apaisée de la conversation civique et de la décision publique. C'est à ce prix que l'on réconciliera l'économie mondialisée avec la promesse démocratique et la sobriété écologique. Partagez-vous cette ambition, madame la secrétaire madame la ministre

Le second, Emmanuel Nizard, atteint du Covid-19, s'est rendu compte qu'il était impossible de se procurer des masques en France. Il s'est donc décidé à changer de métier et à devenir lui-même fabricant. Aujourd'hui, à Meudon, dans une

Cette crise a souligné des carences : pénurie de masques, incapacité de tester massivement les populations, dysfonctionnements dans la chaîne de commandement entre les agences régionales de santé et les préfectures, appels dans l'urgence aux collectivités territoriales. Néanmoins, nous pouvons être fiers du sens civique manifesté par les Français et de l'esprit de responsabilité des élus locaux. Notre République, lorsqu'elle traverse des crises ou est prise de convulsions, a toujours su puiser dans ses ressources pour en ressortir plus forte. Si nos institutions ont été et demeurent solides, l'esprit qui les fait vivre doit être renouvelé. Le pacte social qui nous maintient unis malgré nos différences ne peut plus fonctionner avec les recettes d'hier.

qui ne peut plus être vu comme un reste de l'ancien monde. Ce dialogue, comme l'activité du Parlement, est non pas un obstacle aux réformes et à leur rapidité, mais un passage utile et obligé pour que les réformes proposées puissent être enrichies et marquées d'une légitimité plus grande.

cela veut dire oser le débat, souffrir la contradiction, reconnaître avec humilité que l'on s'est trompé et préférer à la disruption jupitérienne la concorde républicaine, socle incontournable de la reconstruction de notre pays, pour autant qu'elle soit le fruit d'un pacte de confiance scellé au préalable.

propos des allocations familiales. Nous sommes au moins d'accord sur le fait qu'il faut un système de protection sociale fort pour protéger les plus fragiles.

pour une durée que nous espérons définitive, votre réforme du système d'assurance vieillesse, que vous estimiez trop généreux et que vous avez si souvent discrédité depuis trois ans.

paient la crise sanitaire, ce sont les intermittents du travail. Pour eux, le chômage sera plus douloureux. On vous a demandé à plusieurs reprises d'anticiper les effets de la pauvreté.

pour leur garantir un revenu minimum d'existence, un « RSA jeune », quelque chose qui soit plus que la garantie jeunes, mais pas non plus la prime d'activité, qui n'est pas adaptée à des jeunes qui sont intermittents. Enfin, la crise nous l'a appris, le travail au noir est

La séance est reprise. Mes chers collègues, par courrier en date de ce jour, M. Jean-Claude Requier, président du groupe du RDSE, demande que la proposition de résolution visant à encourager le développement de l'assurance de l'assurance récolte, initialement inscrite à l'ordre du jour de l'espace réservé à son groupe du 28 mai, soit inscrite à l'ordre du jour de l'espace réservé à son groupe du mercredi 24 juin, en remplacement du débat sur le thème : « La crise du Covid-19 révélatrice d'un besoin renforcé de déconcentration et de décentralisation ».

dans l'intérêt du dialogue social auquel le mécanisme d'intéressement concourt. L'amendement

pour cette catégorie d'entreprises a vocation à inciter celles-ci à conclure, au terme de trois ans, un contrat d'intéressement dans des conditions classiques. Quel est l'avis de la commission

porte sur l'interdiction de la reconduction tacite d'un dispositif d'intéressement mis en place par voie unilatérale. Comme le Sénat l'avait fait en mars dernier, la commission a souhaité qu'un accord d'intéressement mis en place par voie unilatérale puisse être reconduit tacitement. En effet, la mise en place de dispositifs d'intéressement par voie unilatérale n'est prévue que dans le cas où l'entreprise serait dépourvue de délégués syndicaux à même de négocier un accord. Les choses ont évolué, puisqu'il s'agissait des entreprises de moins de onze salariés. Si, au terme des trois ans de validité du dispositif, l'employeur ne dispose toujours pas d'interlocuteurs de négociation, il serait dommage d'interdire la reconduction de la mesure. Cet amendement me semble donc contraire à l'objectif visé, à savoir favoriser le développement des accords et de la discussion. C'est la raison pour laquelle nous avions émis un avis défavorable.

Il est vrai que le Sénat a déjà eu l'occasion d'adopter un amendement identique, mais la commission des affaires sociales est toujours réticente face à la création de niches sociales et fiscales dont l'impact pour les finances publiques n'a pas été mesuré en amont. En effet, contrairement à la prime exceptionnelle, les sommes versées au titre de l'intéressement sont, comme tous les revenus, assujetties à la CSG, à la CRDS et à l'impôt sur le revenu. Il me semble qu'un dispositif d'exonération totale ne doit être qu'exceptionnel, sous peine de créer un précédent dangereux, voire de traiter de manière inéquitable les salariés en fonction de la taille de leur entreprise. J'ajoute que la difficulté, pour les employeurs qui souhaitent proposer des dispositifs d'intéressement, est grandement réduite par la publication d'accords types mis à disposition par l'administration.

Lubin. Cet amendement vise à limiter la mise à disposition à titre gratuit des agents territoriaux ou hospitaliers auprès des établissements de santé, hôpitaux, établissements médico-sociaux, établissements d'hébergement pour personnes âgées

hospitalière et territoriale au bénéfice des établissements de santé et médico-sociaux, pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, a tout son sens dans ce projet de loi d'urgence. Elle a, dans un objectif de clarté et d'efficacité, été inscrite dans ce texte. Toutefois, la commission a étendu cette dérogation au-delà de la durée de l'état d'urgence sanitaire. Une telle modification permanente devrait impliquer un dialogue avec les instances représentatives et les collectivités. D'ailleurs, la réflexion plus générale sur l'organisation hospitalière que cette pérennisation appelle

se fait sur la base du volontariat entre les hôpitaux et les collectivités territoriales ; en aucun cas ces dernières ne seront dans l'obligation de mettre leurs personnels à disposition pour pallier une quelconque défaillance de l'État. Je rappelle aussi que ce dispositif n'est pas

cette possibilité à la période de l'urgence sanitaire. La dérogation à l'obligation de remboursement en cas de mise à disposition d'agents des fonctions publiques hospitalière et territoriale est destinée à faciliter le renfort des établissements pendant une situation d'état d'urgence sanitaire ; elle ne peut être considérée comme un moyen permanent de renforcer les effectifs de ces établissements. Pour cette raison, le Gouvernement est favorable au rétablissement de la version initiale du texte, qui limitait la possibilité de déroger à l'obligation de remboursement aux seules situations d'urgence sanitaire. Avis favorable, donc, sur l'amendement n° 103 rectifié

de vote. Les maires et les responsables de nos collectivités locales se sont très fortement investis pendant

du bornage dans le temps de cette disposition et celui de la gratuité de la mise à disposition. Je n'imagine guère les élus locaux, demain, accepter de mettre à disposition sans demander le remboursement. Si l'État peut se permettre de le faire,

Dans le cadre de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions a été voté et mis en oeuvre un dispositif de santé publique de gestion des malades du Covid-19 et de leurs cas contacts autour de « brigades de leurs cas contacts autour de « brigades sanitaires ». Les campagnes de dépistage doivent relever de ce dispositif, y compris lorsqu'il s'agit de contamination en milieu professionnel. Cela a été le cas tout récemment, dans des établissements scolaires par exemple. Il n'y a donc pas lieu, à nos yeux, d'étendre la faculté de procéder à des tests de dépistage du Covid-19 aux médecins de prévention de la fonction publique, d'autant que l'objet de cet amendement adopté en commission et devenu article 1 AA justifiait cette extension par référence à ce qui a été prévu pour les médecins du travail. Or le Gouvernement a finalement annoncé que ces derniers ne pourraient y procéder, puisque les campagnes de dépistage sont interdites en entreprise. Le décret d'application de l'ordonnance n'a donc pas rendu effective cette faculté pourtant ouverte par ordonnance. Le Gouvernement a dû faire machine arrière, du fait du risque de non-respect du secret médical. Rien ne justifie donc le dépistage du Covid-19 par les médecins de prévention de la fonction publique. Les fonctionnaires doivent relever du droit commun et d'un dépistage par le système de santé publique.

des agents qui pourraient vouloir se faire tester, ce qui paraît tout à fait légitime. On comprendrait mal pourquoi le corps médical dans son entier, quel que soit son statut, ne serait pas mobilisé. J'émets donc évidemment, au nom de la commission, un avis défavorable sur cet amendement. Quel est l'avis

Ce dispositif a été adopté afin de régler la participation des médecins du travail au dépistage du Covid-19, dans un contexte qui couvre la fonction publique hospitalière et qui, à ce titre, appelait des aménagements. Un ensemble de mesures a ainsi été élaboré, prévoyant d'encadrer les pratiques de dépistage, qui ne peuvent être mises en oeuvre sans un protocole précis. Il est à noter que les dispositions de cette ordonnance sur la question des dépistages sont temporaires et applicables jusqu'au 31 août 2020 au plus tard. Cette approche s'explique par la nature même des tests, les tests virologiques constituant des gestes invasifs très techniques et difficilement réalisables dans le cadre de la médecine du travail et les tests sérologiques n'ayant pas été retenus dans la stratégie nationale

Laurence Cohen, sur l'article. Nous allons voter cet article, qui émane d'un amendement du Gouvernement déposé à l'Assemblée nationale. Autant nous avons quelques doutes sur le caractère urgent de certaines mesures contenues dans ce projet de loi, autant, en l'espèce, il s'agit effectivement d'une urgence, qui aurait d'ailleurs pu faire d'anticipation. Cet article porte sur les maisons de naissance, plus précisément sur la prolongation de leur expérimentation, puisque celle-ci arrive à son terme le 23 novembre prochain.

demandé que ces structures puissent être pérennisées. Tel est également le sens de la proposition de loi de notre collègue Bernard Jomier, qui devait être examinée le 3 juin par la Haute Assemblée. Comme vous le savez, une maison de naissance est un lieu d'accueil et de suivi de grossesse et d'accouchement

pendant le travail ont accouché par voie basse spontanée ; seules 3 % d'entre elles ont eu une césarienne, 3,3 % une épisiotomie, et moins de 3 % une rupture artificielle de la poche des elles ont pu s'hydrater. On le voit : ces données reflètent un certain confort pour les femmes, ce qui n'est pas à négliger, eu égard notamment à certaines pratiques gynécologiques et obstétricales qui sont aujourd'hui de plus en plus considérées comme des violences, et donc dénoncées comme telles. C'est pourquoi nous voterons cet article qui prolonge d'un an leur existence, en attendant un texte plus complet pour préciser le rôle de ces maisons de naissance et proposer leur généralisation sur le territoire. L'amendement Comme vient de le dire très bien à l'instant notre collègue Laurence Cohen, les maisons de naissance ont un bilan positif pour les mères, pour les pères et aussi, semble-t-il, pour les bébés qui y naissent.

reporte en quelque sorte la discussion de fond sur la période post-expérimentation. Nous nous réjouissons que le Gouvernement ait décidé de prolonger l'expérimentation. Pour autant, un petit amendement me semble nécessaire. Il était prévu que le Gouvernement remette au Parlement un rapport d'évaluation un an avant la fin de l'expérimentation,

une nouvelle fois la parole au nom de mes collègues de la commission des affaires sociales. Les laboratoires de biologie médicale sont très mobilisés, dans le cadre de la crise sanitaire, pour la réalisation de tests de dépistage. Or une ordonnance du 13 janvier 2010 avait prévu qu'à compter du 1 novembre 2020 les laboratoires de biologie médicale ne pourraient fonctionner sans disposer d'une accréditation portant sur la totalité des examens de biologie médicale. Du fait de leur activité particulièrement dense dans la lutte contre l'épidémie, il est à craindre que ces laboratoires ne soient pas en capacité de satisfaire à cette obligation dans de tels délais. Il est prévisible qu'ils ne seront pas non plus en mesure de déposer leurs dossiers d'accréditation au 31 octobre 2020, obligation prévue par le projet de loi d'accélération et de

Les laboratoires de biologie médicale sont en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, la stratégie de tests étant montée en puissance avec le déconfinement. Il est apparu sage à la commission, dans ce contexte de crise sanitaire,

elle aurait mérité, peut-être, un examen plus approfondi que ce que permet l'examen de ce projet de loi d'urgence. De surcroît, certaines modalités de cette procédure essentielle pour la qualité et la rigueur des examens de biologie médicale sont renvoyées à un arrêté- c'est le II de Il serait utile que le Gouvernement puisse nous confirmer que l'évolution proposée est bien conforme à ses échanges en cours avec les biologistes et aux orientations souhaitées par la profession.

de biologie médicale, dans le prolongement de dispositions- vous l'avez fort justement rappelé -votées ici même au Sénat. Cet amendement vise à préciser les modalités de mise en oeuvre de l'accréditation définitive des laboratoires de biologie médicale déjà accrédités à au moins 50 des examens de biologie médicale qu'ils réalisent. Compte tenu des efforts déjà consentis par les laboratoires en activité pour atteindre le plus haut niveau possible de qualité, il s'agit de simplifier le processus d'accréditation sans pour autant mettre en cause la qualité et la fiabilité des examens de biologie médicale.

de détresse psychosociale et retarde d'autant plus leur prise en charge. C'est pourquoi le critère psychosocial doit être pris en compte et ajouté à la définition de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique

évoluer les critères de définition même des IMG ; nous serions ainsi au plus près de la réalité vécue par ces femmes et de leurs besoins. Il est

est dépassé- nous reviendrons à l'occasion de l'amendement suivant sur la question du délai légal -, il est possible de recourir à une interruption dite médicale de grossesse quand la santé de l'enfant à naître ou la santé de la mère sont en danger. L'interprétation faite par les équipes médicales de cette disposition relative à l'interruption médicale de grossesse a conduit à élargir la question de la santé de la mère à ce qu'on appelle la détresse psychosociale. Pour faire simple, il s'agit de cas de viols, d'incestes, de femmes handicapées mentales, de situations d'extrême précarité ou de désespoir :

aux médecins d'utiliser l'interruption médicale de grossesse pour répondre aux situations liées aux reports d'IVG pendant la crise sanitaire. dans le collège d'un médecin de médecine foetale, qui n'a pas de raison d'être dans des cas où la question est uniquement celle de la détresse psychosociale de la mère, alourdit considérablement la prise de décision. La collégialité a tout son sens lorsqu'il s'agit d'une interruption réellement

les IMG pour motifs de détresse psychosociale. Il convient de rappeler que les gynécologues-obstétriciens exerçant exerçant en centre de diagnostic prénatal ont l'habitude de traiter des demandes d'IMG pour détresse psychosociale. Il n'y a donc pas lieu de les exclure de cet examen. D'ailleurs le Collège national des gynécologues et obstétriciens français a lui-même lui-même insisté en octobre 2019 sur la nécessité de prendre en compte l'expertise des centres de diagnostic prénatal sur l'IMG psychosociale, cette expertise ne se limitant pas à la seule médecine foetale. Enfin, la modification proposée au travers de l'amendement n° 211 rectifié aurait un caractère non pas temporaire et limité à l'épidémie, mais permanent puisqu'il tend à modifier directement l'article du code de la santé publique régissant les conditions d'examen des demandes d'interruption médicale de grossesse.

entre les deux, le second ne pouvant être le prolongement du premier. Si j'en comprends bien le sens, ces amendements sont en faveur non seulement d'une simplification des procédures d'IMG, mais également d'une extension des conditions pour lesquelles il est possible d'y avoir recours. Les évolutions proposées

dit. J'aimerais qu'à l'occasion de ce débat nous puissions réfléchir ensemble au fait que les problèmes psychosociaux, psychologiques et autres des femmes sont aussi des problèmes extrêmement importants à prendre en compte

au Sénat, à avoir tenté de présenter de tels amendements à différentes occasions. Bien souvent, ils sont frappés d'irrecevabilité

pour explication de vote. J'ai un peu de mal à comprendre le raisonnement. Depuis le 23 mars, nous sommes dans un état de dérogation permanente. Nous dérogeons à la dérogation, en général. Et là, sur un cas qui est circonscrit, tout du moins pour ce qui concerne l'amendement n° 53 rectifié,

s'agit d'inscrire une disposition définitive et non pas au titre d'un problème conjoncturel. Par conséquent, on change la nature même de la disposition

Le scrutin est clos.

Mais ce n'est pas du tout l'objet de l'amendement que je défends à cet instant. Cet amendement est totalement circonscrit sur la période de la crise sanitaire, plus trois mois.

pour des raisons simples. D'abord pour des raisons d'enfermement domestique et familial : il n'est pas si facile que ça de se faire une petite autorisation de sortie et d'expliquer à sa famille, surtout quand on est une jeune femme ou une jeune fille, que l'on s'absente non pas pour aller à la boulangerie, mais pour se rendre dans un centre hospitalier afin de

contre les violences intrafamiliales pendant la crise sanitaire. Pardonnez-moi de le dire, mais je suis presque sûre que, quand il y a violence intrafamiliale et violence conjugale contre les femmes, il y a viol également. Ces violences donneront aussi lieu à des grossesses non désirées. surcroît, je l'ai évoqué il y a un instant, l'été n'est pas un bon moment pour l'activité de tous ces services d'orthogénie et d'IVG. Enfin, l'un de nos collègues a évoqué le fait que l'on était en train de sortir de la crise sanitaire.

pendant la période de la crise sanitaire, plus trois mois, est une demande qui émane des médecins. N'obligez pas les médecins à se mettre hors la loi pour répondre à la détresse des femmes ! Il faut entendre ce que nous demandent les médecins.

trois minimum au-delà de la crise sanitaire -, il va falloir assumer des IVG avec un peu de dépassement de délai. C'est pourquoi il serait raisonnable pour nous tous voter ce délai de deux semaines supplémentaires.

et que nous continuons quand même de traverser, les hôpitaux qui pratiquent les IVG ont été conduits à demander aux femmes de ne pas s'y présenter. Ils étaient mobilisés

L'amendement n° 58 rectifié vise à allonger temporairement jusqu'à trois mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire le délai légal pour réaliser une IVG, en le portant de la fin de la douzième semaine de grossesse à la fin de la quatorzième semaine. semaine. Le Gouvernement a déjà mis en place un dispositif pour adapter l'accès des femmes à l'IVG pendant l'épidémie en assouplissant le recours à l'IVG médicamenteuse et en rappelant, pour les recours tardifs à l'IVG instrumentale, la possibilité de recourir à l'IMG pour motif de détresse psychosociale de la femme. Toutefois, la commission a estimé qu'une IMG est une procédure lourde, qui requiert au préalable l'accord de deux médecins, après une concertation pluridisciplinaire. Elle peut prendre du temps, parfois une semaine, voire plus. L'IMG pour motif de détresse psychosociale ne lui est donc pas toujours apparue pertinente pour des femmes confrontées à des difficultés de prise en charge pendant la crise sanitaire. L'amendement visant à un allongement du délai strictement temporaire justifié par le caractère exceptionnel de la crise sanitaire que nous traversons, il ne saurait donner lieu à une remise en cause pérenne du délai légal de l'IVG, qui doit, dans l'absolu, à l'issue de la crise, toujours rester limité à douze semaines de grossesse. Moyennant cette condition, la commission a émis un avis favorable.

de nombreuses activités hospitalières et à conseiller de reporter un certain nombre de soins non urgents, le cas échéant. Dans ce contexte, nous avons craint des difficultés d'accès à l'avortement ; c'est le retour que nous ont fait un certain nombre de professionnels de santé et les associations comme le planning familial. Ici même, sur ces travées, et à l'Assemblée nationale les parlementaires se sont fait le relais de ces craintes et de ces difficultés. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a agi très rapidement et très fortement, de façon dérogatoire, le temps de l'urgence sanitaire. Nous avons permis la réalisation de l'ensemble des consultations obligatoires sous forme de télémédecine, la consultation de prise des pilules contraceptives, ce qui a nécessité de changer le circuit du médicament, désormais accessible en pharmacie. Pour garantir le secret des avortements pour les jeunes filles mineures, nous avons modifié les attestations de déplacement en période de confinement pour que n'y figure plus l'autorisation parentale. Pour davantage simplifier les démarches, le ministre des solidarités et de la santé a demandé à la Haute Autorité de santé si nous ne pouvions pas allonger la période durant laquelle il était possible de réaliser un avortement médicamenteux hors hôpital.

Le 14 avril, soit quatre jours plus tard, nous avons pris un arrêté allongeant le délai de l'avortement médicamenteux réalisable à domicile. J'entends que certains veulent aller plus loin dans cette période de crise et allonger le délai de l'IVG, mais le Gouvernement n'y est pas favorable. C'est un débat que vous avez déjà mené dans cet hémicycle, mais qui est beaucoup plus global. Il ne nous paraît pas en adéquation avec les mesures que nous avons essayé de prendre et qui ont été prises formellement pour tenter de résoudre la situation d'un certain nombre de

S'agissant de rendre la mesure applicable jusqu'à trois mois après l'état d'urgence sanitaire, dans l'hypothèse où l'état d'urgence sanitaire se limiterait au 10 juillet, nous sommes en train de parler d'enfants qui ne sont pas encore conçus. Cela signifie que nous visons un public qui n'est pas celui qui a été atteint par le confinement. Nous savons donc pertinemment que si nous mettons un tel délai en place nous ne pourrons jamais revenir en arrière.

Est-ce cela que nous attendons du débat démocratique ? Je ne le crois pas ! Passer de douze à quatorze semaines de grossesse pour le délai d'IVG n'est pas une décision anodine,

Comment trouver un système

l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Le récent bilan de l'application des lois établi par la commission des affaires sociales a fait état d'un faible taux d'application de cette loi, monsieur le ministre : 30 % au 31 mars 2020, soit six mois après sa promulgation, sa promulgation, et aucune des onze ordonnances prévues n'a été publiée. Force est de constater que la crise sanitaire ne constitue pas, depuis le début de l'année, un contexte propice à l'avancée des concertations et des travaux sur de nombreux sujets.